La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

début de cette année, après les arbitrages, le projet de loi a été présenté au Conseil d'État, qui a émis, comme on le dirait au Quai d'Orsay, un avis « mesuré et réservé

? La parole est à M. le Premier ministre. Monsieur le président Marseille, comme vous l'avez rappelé, le Président de la République s'est engagé, au moment de son élection, à mettre en oeuvre une réforme majeure consistant à refonder notre pacte social, afin d'installer un système universel de retraite.

suscitent des oppositions, des contradictions, des débats, des questionnements. Pour connaître comme moi la vie politique française et le débat public, vous savez que toucher aux retraites, c'est faire naître ces questionnements, ces critiques, ces oppositions et, parfois, il est vrai, des manifestations ou des blocages.

étude d'impact, qui, vous le savez, comptait près d'un millier de pages. Je suis certain que tout le monde s'est engagé dans cette lecture

Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il permettra d'élaborer un texte encore meilleur que celui que nous soumettons au Parlement, car c'est à cela que sert l'examen parlementaire. Cependant, je veux être clair, monsieur Marseille

Monsieur le Premier ministre, ni triomphalisme ni relâchement : le chômage est la plus grande injustice sociale de notre pays et tout le monde doit contribuer à la lutte. Si le chômage ne vous intéresse pas, dites-le-moi, chers collègues ! J'en préviendrai nos compatriotes Les chiffres publiés cette semaine sont éloquents, avec 120 000 chômeurs de catégorie A de moins sur un an, soit la plus forte baisse enregistrée depuis 2007. La réforme du code du travail, de l'apprentissage, de la formation continue, les baisses de charges et d'autres mesures prises par le passé n'y sont pas étrangères.

car, si les chiffres montrent que la croissance, bien que modérée, est créatrice d'emplois, notamment de CDI, ce constat ne doit pas nous dispenser d'une grande exigence quant aux chantiers que nous avons à mener tous ensemble : grand plan de formation pour les chômeurs de longue durée ou les jeunes sans qualification, augmentation du taux d'emploi des seniors, comme le préconise le rapport Bellon, réponse au cas des nombreuses offres d'emploi non satisfaites Premier ministre, ma question est simple : comment le Gouvernement entend-il poursuivre la lutte contre le chômage qu'il a entamée et quelles sont les mesures qui seront prises dans les mois à venir pour parvenir à ce que l'injustice que constitue le chômage régresse dans notre pays ? La parole

j'ai souvent pensé que nous avions, en France, une difficulté particulière à nous réjouir collectivement de bonnes nouvelles.

et c'est toujours une bonne nouvelle pour le pays. D'importantes annonces ont été réalisées dans le cadre du sommet organisé par le Président de la République. De ces bonnes nouvelles, je veux me réjouir. Elles ne sont pas évidemment sans lien avec les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. De fait, les chiffres du chômage sont bons. Plus exactement, ils montrent une tendance continue à l'amélioration. Nous devons nous en réjouir, pour ceux qui

qu'il faut corriger. C'est ce que nous essayons de faire, au travers des plans de formation, de la réforme de l'assurance chômage, du développement de l'attractivité de notre territoire et de l'ensemble des mesures fiscales que nous avons prises, que nous assumons et qui- réjouissons-nous-en, mesdames, messieurs les sénateurs -commencent à produire d'excellents effets.

nationale et de la jeunesse, nombre de nos départements ruraux font face à la déprise démographique. La présence d'un bon maillage d'établissements scolaires est un enjeu d'autant plus fondamental qu'il contribue à attirer et à fixer des familles, à faire vivre l'économie locale et à développer de véritables savoir-faire dans nos territoires. L'internat peut constituer une réponse adéquate. Or la désaffection à son égard est bien documentée. En 1960, près d'un quart des élèves du second degré étaient internes. Ils sont moins de 4 % aujourd'hui, alors qu'il existe près de 40 000 places vacantes. Monsieur le ministre, vous avez décidé de revitaliser et de moderniser ce modèle d'enseignement. Pour ma part, j'y vois un moyen d'insuffler du dynamisme et de la jeunesse dans des territoires vieillissants. Après la remise du rapport de Jean-Yves Gouttebel et de Marc Foucault, vous avez présenté un plan pour l'internat du XXI siècle, qui a pour ambition de créer ou de rénover 100 internats d'excellence, 100 résidences à thèmes et 40 campus professionnels d'ici à 2022, pour un total de 13 000 places. Ce projet a, en particulier, pour finalité de tisser des liens étroits avec les territoires ruraux. Bien sûr, en tant que sénatrice du Cantal, je m'en réjouis, mais je m'interroge aussi sur l'appel à projets destiné aux collectivités qui a été annoncé pour la rentrée. Quel est son calendrier ? Quelles sont ses modalités ? Plus largement, comment se coordonneront l'État et les collectivités pour atteindre les objectifs, sachant que les territoires qui en ont le plus besoin ne disposent généralement pas des ressources nécessaires ? Enfin, de quelle façon allez-vous articuler ce projet éducatif à celui des campus connectés ? L'ouverture annoncée d'une centaine de sites d'ici à 2022 pourrait, si leur localisation était coordonnée avec le plan pour l'internat, offrir des perspectives nouvelles pour nos territoires. La parole

fermeté. Votre question est très importante, parce qu'elle porte sur l'une des politiques publiques les plus importantes qui puissent être en matière sociale et en matière d'aménagement du territoire, comme vous l'avez très bien dit.

citoyen et écologiste. Monsieur le Premier ministre, avec votre texte sur la réforme des retraites, vous faites preuve d'un triple mépris. Mépris du peuple, qui, majoritairement, continue de s'y opposer. Mépris du Parlement,

aux gouvernements futurs de suivre votre politique. Décidément, le respect du peuple et des institutions n'est pas votre credo ! En vous attaquant ainsi à ces retraites voulues par le Conseil national de la Résistance, font aujourd'hui République et contribuent au pacte social, vous fragilisez durablement ce que sera, demain, notre société. Oui, monsieur le Premier ministre, je vous le redemande : quand allez-vous retirer ce projet dangereux, anticonstitutionnel et encore aujourd'hui très

de l'engagement démocratique pris par une majorité de députés devant tous leurs électeurs ? Voilà un témoignage du respect de la démocratie.

la sénatrice, sur le fait que nous ne retirerons pas notre projet de loi et que nous nous honorerons de le porter jusqu'au bout

dit la population. Il faut entendre les évolutions de la société ! Or force est de constater qu'aujourd'hui, au bout de deux ans et demi, vous avez accumulé plus de colère sociale qu'il n'y en a eu sous les quinquennats de Nicolas Sarkozy et François Hollande réunis. Est-ce pour vous un gage de réussite En faisant cela, vous continuez de fragiliser notre République. Vous serez, demain, les responsables du chaos démocratique dans notre pays !

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, manque de temps, complexité des textes, modifications en cours de route, projections financières lacunaires, étude d'impact insuffisante, insécurité juridique

qui plus est dans le contexte de relative solidité auquel ont abouti les réformes successives. En outre, le renvoi à 29 ordonnances sur des sujets majeurs interdit une vision globale. Hier, à l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre a admis qu'une refonte aussi complète, fondée sur des hypothèses économiques étant toutes susceptibles de bouger, pose beaucoup de questions. Là, nous sommes tous d'accord. Bienvenue au club ! Ma question est simple engager une procédure accélérée sur un tel texte, alors qu'il s'agit d'une réforme systémique, contrairement aux réformes précédentes ? Pourquoi déconnecter la conférence de financement de l'examen parlementaire ?

... Le Conseil d'État s'est exprimé dans son rôle de conseil du Gouvernement. Il l'a très bien fait ! À ce titre, il a donné un certain nombre de conseils au Gouvernement. Le Gouvernement les entend et les prend en compte. Il ne vous a pas échappé que, dans sa note de 63 pages, le Conseil d'État a également validé la quasi-totalité des dispositions des deux projets de loi, notamment leurs dispositions tendant au respect de normes internationales à l'égard desquelles nous sommes engagés, mais également de dispositions constitutionnelles.

la réplique. Très sincèrement, quel gâchis ! Nous sommes pourtant dans une période propice pour réformer sur le fond, puisque le système est quasiment sécurisé jusqu'en 2030. Il permet de poser des questions de fond incontournables : augmentation de l'espérance de vie et du nombre des seniors, lacunes de notre système face aux mutations économiques et sociologiques, problèmes des femmes, carrières hachées, inégalités d'espérance de vie, pénibilité, nécessaire recherche de nouveaux modes de financement ... Ce projet n'est pas un projet de retraite universel. C'est simplement un système universel par points. C'est un projet qui ne répond pas aux inégalités. Pis, il peut les aggraver En bref, à l'insécurité juridique s'ajoute, aujourd'hui, l'insécurité sociale.

ces chiffres sont connus et inquiètent, à deux jours du Brexit. La rencontre de la semaine dernière entre le président de la région Bretagne et le commissaire en charge de ces sujets en est une preuve, tout comme les alertes des pêcheurs de toute la façade maritime de Dunkerque à Brest. La pêche représente moins de 0,1 % du PIB du Royaume-Uni. Pourtant, le contrôle des eaux de pêche et leur ouverture furent l'un des points de crispation des discussions outre-Manche avant le référendum. Le poids politique est donc sans commune mesure. Boris Johnson l'a bien compris. La pêche sera ainsi un axe phare des négociations houleuses du Brexit. Les interrogations sont nombreuses, dans le Nord comme ailleurs. Elles portent sur l'accès aux eaux britanniques après décembre 2020, mais aussi sur la concurrence induite par la possible réorientation des flux de pêcheurs européens vers notre espace maritime. Les États membres vont prochainement donner mandat à la Commission européenne pour négocier la relation future avec le Royaume-Uni. Pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, nous assurer que la filière pêche ne se retrouvera pas emprisonnée dans un statut de variable d'ajustement face à un accord économique plus complet ? Pouvez-vous également nous éclairer sur les mesures relatives au secteur de la pêche que la France et l'Union européenne ont prévues pour faire face à une éventuelle absence d'accord, finalement toujours d'actualité

mais les pêcheurs, eux, ne quitteront pas les eaux britanniques. Comme vous l'avez rappelé, ils auront accès à ces eaux au moins jusqu'au 31 décembre 2020. Les Britanniques continueront d'appliquer pleinement les règles de la politique commune de la pêche jusqu'à

Les mesures étaient prises pour le cas où il n'y aurait pas eu d'accord le 31 janvier. Des fonds seront disponibles en cas de cessations d'activité. Ce n'est pas notre scénario et je préfère, dans les mois qui viennent, travailler avec vous

des enseignants, des policiers et des pompiers, les avocats qui mettent leur robe à terre, ports bloqués, manifestations syndicales à répétition, entreprises en difficulté, une économie lourdement touchée, des commerçants qui n'en peuvent plus, ajoutez à cela une réforme des retraites conduite avec un incroyable amateurisme qui a suscité de grandes inquiétudes chez nos concitoyens Face à ces inquiétudes, votre majorité a fait preuve d'une grande arrogance et d'une cacophonie anxiogène. Le résultat est là depuis quatorze mois : la chienlit est installée et les Français ont perdu confiance. Monsieur le Premier ministre, quand et comment comptez-vous ramener la confiance et la sérénité dans notre pays qui en a tant besoin ?

nous nous sommes engagés dans des transformations dont j'ai parfaitement conscience qu'elles suscitent des réactions, des questionnements, des angoisses, parfois des oppositions très fortes, mais auxquelles il était

alors que le Président de la République a récemment évoqué les problèmes que posent le communautarisme et le séparatisme islamistes, sans indiquer comment il compte les combattre, une adolescente de 16 ans fait face, quasiment seule, à une vague de haine et de violence sans précédent et n'est plus scolarisée. En effet, pour le seul crime d'avoir critiqué une religion, l'islam, après avoir été harcelée sur les réseaux sociaux, la jeune Mila est aujourd'hui victime de ce qui peut être comparé à une, confortée par la prise de position honteuse et inadmissible du délégué général du CFCM,

ont critiqué l'islam. Entre les insultes homophobes et les menaces de mort, Mila est devenue en quelques jours le symbole de la volonté des islamistes d'anéantir notre liberté d'opinion et d'expression et de réinstaurer le délit de blasphème en France. Il n'y a pas de racisme dans le fait de critiquer une religion, quelle qu'elle soit. L'islam, comme toutes les autres religions, doit se soumettre à la critique, à l'humour et aux lois de la République. Monsieur le Premier ministre, musulmane pour l'islam de France, dans laquelle les Frères musulmans sont très présents, eux qui remettent systématiquement en cause notre liberté de conscience et d'expression, le Président de la République parviendra-t-il à imposer à certains musulmans qui ne veulent pas l'entendre notre droit de critiquer toutes les religions

le faire. Il est inacceptable, insupportable même, que certains, au nom de l'institution qu'ils représentent, aient pu laisser penser que cela était interdit. Nous devons,

Monsieur le ministre, dans une France plus fracturée que jamais, dans un climat d'inquiétude et de peur, les propos de Mme la garde des sceaux ce matin, à la radio, ne font que conforter mes doutes et mes interrogations. Non, madame Belloubet, injurier et critiquer une religion n'est pas une atteinte à la liberté de conscience.

les États-Unis de Donald Trump ont décidé d'augmenter les taxes à l'importation sur une liste de produits européens. Parmi eux, une fierté nationale et le deuxième contributeur aux exportations du pays : le vin. J'englobe bien évidemment dans ce secteur les productions de Bourgogne, où l'on a fêté la Saint-Vincent ce week-end, mais c'est bien l'ensemble de la production nationale qui est concerné : les vins de Bordeaux, de l'Hérault, de Champagne, les vins de Gascogne, le chablis, les vins de la Drôme et même l'irouléguy, une AOC très appréciée à Biarritz Ces produits souffrent d'une surtaxation de 25 % depuis octobre dernier sur le marché américain. La filière craint les effets de cette guerre commerciale sur le long terme. Elle s'interroge sur la durée du maintien de cette surtaxe. Et nous savons tous qu'une part de marché perdue met des années à être regagnée. On nous dit que le climat commercial avec M. Trump pourrait changer en raison de décisions de justice à venir dans le secteur de l'aéronautique. On nous annonce aussi une paix des braves sur le front des GAFA. Mais la viticulture française attend des réponses concrètes et rapides. Elle demande la constitution d'un fonds de 300 millions d'euros. En octobre dernier, le ministre de l'agriculture annonçait avoir demandé à l'Union européenne « de prendre des mesures d'accompagnement pour faire face à cette situation exceptionnelle ». Le Gouvernement pourrait-il nous indiquer ce que le ministre a obtenu avant de tourner son attention vers les Pyrénées-Atlantiques ? Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous n'aurez que la réponse d'un ancien ministre de l'agriculture, ... Et de droite ! ... mais j'espère qu'elle vous conviendra.

La parole est à M. Jacques Grosperrin, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le bilan de la délinquance en 2019 est mauvais tous les indicateurs publiés discrètement par le ministère de l'intérieur sont au rouge. Il est loin le temps où le ministre présentait les résultats de son action devant la presse ! À la lecture des chiffres, on comprend cette humilité nouvelle

La police de sécurité du quotidien n'a pas inversé la tendance. Dans mon département, voilà deux ans, le ministre de l'intérieur était venu installer la police de sécurité du quotidien dans Nous allions voir ce que nous allions voir, le Gouvernement avait trouvé la solution, nous disait-on. Ce que nous avons vu, avec un commissariat ouvert à dix heures et fermé à dix-sept heures, ce sont des tirs de balles journaliers, huit blessés à ce jour, une fourrière incendiée avec plus de 160 véhicules, une grande surface hors d'état La réponse pénale est si faible qu'elle assume une forme d'impunité désespérant trop souvent les forces de police. Pensez-vous, monsieur le Premier ministre que la politique annoncée et assumée par la garde des sceaux

Nous devons mener un combat inlassable sur ces sujets. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé un programme de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. C'est la raison pour laquelle, dans 47 quartiers de reconquête républicaine (QRR), nous mettons en place des moyens spécifiques. C'est la raison pour laquelle, parce qu'il faut avoir confiance dans notre police, mais aussi parce qu'il faut lui donner les moyens d'agir, engagé un programme de paiement des heures supplémentaires dont certaines remontent à 2005. C'est aussi la raison pour laquelle nous expérimentons de nouveaux cycles d'horaires de travail, pour plus de présence sur le terrain. Monsieur le sénateur,

pour faire en sorte que chaque mètre carré de la Planoise, de Besançon et de l'ensemble du territoire national soit mieux sécurisé. C'est ce que nous devons à l'ensemble des Français, c'est ce que nous devons aussi aux habitants de la Planoise. C'est le sens d'un budget, monsieur le sénateur,

une remise en cause des choix opérés depuis le début du quinquennat est non seulement une impérieuse nécessité, mais surtout une urgence absolue pour l'autorité de l'État. La parole est à Mme Dominique Vérien, pour le groupe Union Centriste.

Depuis l'annonce de la réforme des retraites qui a provoqué la grève des avocats, les tribunaux dysfonctionnent partout en France. Or, en matière pénale, et plus particulièrement pour les personnes dont la détention provisoire ou la garde à vue arrive à son terme, l'urgence est là. Que faire ? Remettre en liberté des personnes potentiellement dangereuses dans l'attente d'un jugement ? Les juger sans avocat, comme le permet la jurisprudence de la Cour de cassation ? Aucune de ces deux solutions n'est acceptable. Il vous faut donc sortir de la crise. Deux réformes de la justice sont prévues, l'une en mars, sur les peines, l'autre en octobre, sur la justice pénale des mineurs.

éprouvent des difficultés financières, notamment en fin de carrière. Le Gouvernement s'est également engagé à limiter l'impact des hausses de cotisations sur les cabinets, notamment avec la pérennisation de l'abattement permettant de compenser l'augmentation des cotisations

service public de la justice fonctionne dans de bonnes conditions. Le Gouvernement reste ouvert au dialogue, mais dans le cadre qui a été fixé, celui d'un système universel de retraite où chaque Français cotisera à une seule et même caisse.

ampleur. De nombreuses productions conchylicoles sont touchées : en Méditerranée, dans la Manche, sur la côte atlantique ... Dans le Morbihan, deux entreprises sur trois ont dû fermer.

Les pluies abondantes intervenues en fin d'année et au début de cette année, associées aux épidémies hivernales et à une forte consommation d'huîtres, ont très probablement contribué à la survenue de ces infections. La fermeture des zones de production concernées montre la réactivité des services de l'État pour protéger les consommateurs. La vigilance dont fait l'objet la filière est aussi une garantie de qualité des produits mis sur le marché. Toutefois, comme vous l'avez souligné, ces fermetures ont des conséquences économiques et sociales importantes pour la filière. Les responsables ont en effet été reçus au ministère de l'agriculture, et les préfets sont en train de recenser, d'identifier cas par cas les préjudices subis par les entreprises dans les zones concernées. Même s'il ne s'agit pas du seul facteur, cet incident montre l'importance pour les collectivités locales de maîtriser l'assainissement des eaux usées, y compris lors des épisodes de fortes pluies. Le contrôle des rejets des stations d'épuration, des réseaux d'eaux pluviales et des épandages dans les zones conchylicoles font partie des priorités du contrôle, les agences de l'eau apportant par ailleurs des aides aux collectivités pour financer les traitements renforcés des eaux usées, qui sont nécessaires dans ces zones fragiles. Je le rappelle, dans le cadre du onzième programme d'intervention des agences de l'eau, 3,6 milliards d'euros d'aides sont accordés au titre du traitement des eaux usées. Il faut traiter les situations des entreprises en urgence et, globalement,

Concernant plus particulièrement la relation commerciale, qui constitue probablement l'aspect le plus important, le Premier ministre britannique a indiqué que son objectif était de faire du Royaume-Uni une zone d'attrait économique, soit une sorte de Singapour européen, à vingt kilomètres de nos côtes.

à l'égard de l'Union européenne. Le Parlement européen en débat en ce moment, et le Conseil devrait valider formellement, aujourd'hui, l'accord de retrait. Observons d'abord que cet accord de retrait a évité une sortie désordonnée que nous craignions auparavant.

l'autonomie de décision de l'Union européenne et l'équilibre entre les droits et les obligations. Troisièmement, nous ferons en sorte de toujours privilégier le fond sur le calendrier. Il ne faudrait pas que l'urgence se transforme en précipitation

Il est parti ! Monsieur le ministre, le 19 décembre dernier, à quelques jours de Noël, le Président de la République s'adressait à la communauté française

Monsieur le ministre, comme ces millions de Français qui ont entendu ces promesses à quelques jours de Noël, je n'ai pas été vraiment surpris de voir qu'il n'y avait rien, le 25 décembre, au pied du sapin. Il n'y avait rien, alors que, depuis 2013 et les premières fermetures arbitraires de comptes, la situation n'a cessé de se détériorer. Il n'y avait rien, alors que, à chacun de mes déplacements à l'étranger, je suis interpellé par ces Français, qui me font part de leur désarroi et de leur incompréhension. Monsieur le ministre, est-il normal que ces Français soient contraints de se tourner vers des banques étrangères pour ouvrir un compte ou chercher des financements ? Cette situation inacceptable n'a que trop duré. Les Français de l'étranger sont fatigués d'entendre toujours les mêmes promesses. Ils ne supportent plus cette stigmatisation, ils ne supportent plus d'être une variable d'ajustement, de voir leur fiscalité augmenter pendant que les services consulaires voient peu à peu leurs moyens diminuer.

allez-vous enfin exaucer le voeu des Français de l'étranger en luttant réellement contre les pratiques de débancarisation, comme vous l'a demandé le Président de la République ?

dans le code monétaire et financier un droit au compte. Certes, les conditions de résiliation des comptes ont été encadrées. Mais nous constatons que, dans la réalité, un certain nombre d'établissements bancaires font de la surconformité par rapport à des réglementations de lutte contre le blanchiment ou le terrorisme. Ainsi, un certain nombre de nos compatriotes, qui sont pourtant de bonne foi, souvent établis depuis des décennies partout dans le monde, se voient fermer leur compte de façon arbitraire. Face à une telle situation, nous souhaitons, avec Bruno Le Maire, avancer rapidement. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que,

de trouver des solutions concrètes. Tout comme vous, je tiens des permanences de proximité auprès de nos compatriotes établis hors de France. Il y a également le sujet des certificats de vie. Avec Jean-Yves Le Drian, nous l'avons dit à nos services consulaires, il est important d'apporter des réponses lorsque nos compatriotes se heurtent à des procédures

socialiste et républicain. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Le coronavirus nous donne aujourd'hui un nouvel exemple de la globalisation de notre planète, qui fait qu'une crise sanitaire à l'autre bout du monde nous concerne tous. Les médias et les réseaux sociaux nous informent en continu des décisions prises pour apporter une réponse mondiale à l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait plus de 132 morts et contaminé 6 000 personnes en Chine, si je me réfère aux chiffres communiqués ce matin. Chacun s'active pour tenter de contrôler la propagation du virus face à la progression très rapide de l'épidémie, qui touche désormais 14 pays, dont le nôtre. Je souhaite vous interroger, monsieur le ministre, sur les mesures concernant nos compatriotes vivant à l'étranger. La presse annonce le rapatriement de 250 Français et une centaine d'Européens, dont l'avion devait partir ce matin. Mais qu'en est-il des dizaines de milliers d'autres Français vivant en Chine, alors que la France a promis le retour à ses ressortissants qui le souhaitent ? Certains d'entre eux, à Wuhan, nous signalent qu'ils n'arrivent pas à obtenir d'informations sur Qu'en est-il des conjoints chinois ou étrangers qui ont besoin d'un visa pour sortir ? Comment l'obtiennent-ils puisqu'ils ne peuvent se déplacer au consulat ? Aux dires des experts, le pic de l'épidémie devrait être atteint dans une dizaine de jours. L'OMS ne recommandant pas de telles évacuations d'étrangers, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui a motivé votre décision ? nous dire comment sera assuré le suivi de la quarantaine des rapatriés, qui dure quatorze jours, afin de s'assurer qu'elle est bien respectée ? Enfin, comment et où seront traités ceux qui présentent des symptômes suspects et qui seront évacués dans un avion séparé du reste des candidats au départ ? Monsieur le ministre, les questions sont nombreuses. Afin d'éviter l'angoisse et la panique souvent engendrées par l'ignorance, il me semble important de rassurer au maximum nos compatriotes, en les informant régulièrement. Certains estiment d'ailleurs les informations du ministère trop parcellaires. ailleurs, n'oubliez pas les parlementaires représentant les Français établis hors de France ! Nous sommes des relais naturels pour nos compatriotes, qui nous questionnent beaucoup et cherchent auprès de nous des informations fiables. Elles le seraient d'autant plus si elles nous étaient fournies directement par le centre de crise du quai d'Orsay.

je vous remercie de votre question, qui me permet de faire un point sur la situation, laquelle inquiète- c'est bien compréhensible -nombre de nos concitoyens. Le 7 janvier dernier, les autorités sanitaires chinoises ont annoncé la découverte d'un nouveau coronavirus. Le Gouvernement français est depuis pleinement mobilisé afin d'éviter la propagation du du virus sur notre territoire et un suivi quotidien de la situation épidémiologique en France a été mis en place. Comme vous le savez, la situation internationale a évolué, vous en avez rappelé les différents chiffres. En France, un quatrième cas a été confirmé hier. Il s'agit d'un touriste chinois de plus de 80 ans, actuellement hospitalisé. S'agissant du rapatriement et de toutes les questions que vous avez soulevées, un dispositif permettant de rapatrier nos compatriotes est en cours d'organisation, conformément à la demande du Premier ministre. Des contrôles médicaux de préembarquement, réalisés par des équipes spécialisées françaises, permettront d'organiser le retour par avion dans les meilleures conditions de santé publique pour tous. Les modalités précises sur le nombre, la nature des vols et leurs horaires dépendront de la situation et des impératifs de santé publique. Elles n'ont pas vocation à être communiquées à ce jour. Notre objectif est que tous nos compatriotes qui le souhaitent soient assurés de leur retour. Nous faisons le choix de la transparence depuis le début. Le Gouvernement s'engage à continuer ainsi. C'est la seule voie valable, non seulement pour rassurer nos concitoyens, mais aussi pour freiner la propagation du virus. Permettez-moi également de le rappeler, tous les soirs, au ministère, se tient une conférence de presse où l'ensemble de ces sujets sont abordés. Nous apportons les réponses dès lors que nous avons des réponses précises à apporter. La parole

la liste d'aucun groupe. J'aurais pu poser une question à M. le Premier ministre sur ce qu'il pensait des déclarations de son ancien secrétaire d'État Benjamin Griveaux sur l'intérêt du déplacement de la gare de l'Est.

affectent notamment le sud de la France. Vous le savez, nous avons d'ores et déjà un plan national d'adaptation au changement climatique, dont nous avons eu l'occasion de débattre à plusieurs reprises dans cet hémicycle. nous devons manifestement aller plus loin, en particulier pour prendre en compte l'impact de la sécheresse sur les activités de nos agriculteurs, ce qui nous amène à repenser l'ensemble de la gestion du cycle de l'eau. était bien l'objet des Assises de l'eau pilotées, voilà quelques mois, par mon ministère. Elles doivent déboucher sur des réponses très concrètes. C'était notamment le sens de l'instruction qui a été adressée par mon ministère, en lien avec le ministère de l'agriculture, pour inciter à la préparation de programmes de programmes territoriaux pour la gestion de l'eau, dans lesquels les agriculteurs, les industriels, les collectivités et les ONG sont invités à réfléchir ensemble aux besoins et aux économies qui seront nécessaires dans le cadre de la C'est aussi toute la politique de prévention des inondations qui est en cause. J'ai pu m'en rendre compte dans mes déplacements, les élus attendent de nous que nous agissions plus vite en la matière. C'est donc bien un programme d'ensemble que nous devons préparer

La parole est à M. Jean Louis Masson, pour un rappel au règlement. Madame la présidente, l'article 27 de la Constitution dispose : « [ ...] Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. »

Annie Delmont-Koropoulis. Je souhaite faire une mise au point concernant le scrutin public n° 86 : Brigitte Lherbier et Antoine Lefèvre souhaitaient s'abstenir

et de la loi du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- trente et une voix pour, trois voix contre -au renouvellement de M. Philippe Wahl à la présidence du conseil d'administration de La Poste. L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur le contrôle, la régulation et l'évolution des concessions autoroutières. En application de l'article 8, alinéa 5 de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement.

qui introduit la pratique de tests génétiques en première intention dans le cadre du dépistage néonatal. Cet article vise à préciser, en outre, que la prise en charge financière de ces tests serait alors à la charge des titulaires de l'autorité parentale et, éventuellement, des mutuelles complémentaires. Le seul fait qu'un test soit disponible et réalisable ne justifie ni sa prescription ni sa réalisation. La pratique de tests génétiques en première intention dans le cadre du dépistage néonatal doit continuer à répondre aux critères de pertinence des programmes nationaux de dépistage en population générale. Il revient à la Haute Autorité de santé en liaison avec l'Agence de la biomédecine, de travailler sur ces sujets pour étudier les perspectives, notamment thérapeutiques, qui peuvent exister une fois que ces tests ont été réalisés, pour examiner la pertinence de ces tests et pour ouvrir les débats sur des questions qui, à ce stade, ne sont pas expertisées. Le dépistage néonatal a pour objet la prévention secondaire des maladies à forte morbidité ou à forte mortalité dont les manifestations peuvent être prévenues complètement ou partiellement par un traitement engagé très tôt après la naissance. Ce qui justifie c'est l'existence d'un traitement qui peut être commencé immédiatement. Ce dépistage est en France d'excellente qualité, il répond à des besoins précis en santé, sur un public parfaitement identifié, avec des tests validés et performants, et surtout un gain indéniable

Le programme national de dépistage néonatal évolue donc en fonction des avancées scientifiques et des possibilités thérapeutiques. Les examens réalisés dans le cadre de ce dépistage sont fixés par arrêté, en application d'une disposition de principe du code de la santé publique.

du dépistage néonatal. Une fois de plus, je le précise, ce dépistage doit pouvoir conduire à un traitement ou à la proposition d'une thérapie. Un tel article serait source d'inégalités, ce qui n'est pas acceptable. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose d'adopter cet amendement

Certaines maladies génétiques d'une particulière gravité font aujourd'hui l'objet de thérapies géniques prometteuses qui représentent un véritable gain de chances pour les personnes concernées, notamment lorsque ces thérapies sont administrées à un stade précoce chez le jeune enfant, idéalement avant l'apparition des premiers symptômes. C'est le cas en particulier pour certaines formes de l'amyotrophie spinale infantile. Le dépistage de ces maladies nécessite un examen ciblé de génétique moléculaire qui permet d'identifier la présence d'une mutation génétique bien précise. Ce test, peu coûteux, permettrait de faire bénéficier les nouveau-nés concernés par cette mutation de traitements qui amélioreraient significativement leur espérance et leur qualité de vie. À titre d'exemple, il existe un traitement pour une forme de l'amyotrophie spinale infantile qui, s'il est administré très tôt au nouveau-né, permet de prévenir l'apparition de séquelles très lourdes. Toutefois, pour pouvoir procéder à l'injection avant l'apparition des premiers symptômes, il faut savoir si l'enfant présente la mutation génétique en cause. Ce test est envisageable pour un enfant déjà né, il n'y a donc aucune dérive eugénique. Il s'agit, au contraire, de lui permettre d'avoir accès le plus tôt possible aux traitements disponibles.

Or l'AFM-Téléthon nous a indiqué que l'intérêt de ce traitement est qu'il soit administré le plus tôt possible avant l'apparition des premiers symptômes. Les associations de malades demandent donc de pouvoir procéder au test génétique ciblé pour savoir si l'enfant

chez le nouveau-né dans le cadre d'un dépistage néonatal pour la recherche d'anomalies génétiques susceptibles de mesures de prévention. Mme la rapporteure vient de le souligner, des maladies génétiques très graves

D'autres maladies peuvent être recherchées, comme la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie, la mucoviscidose ou la drépanocytose.

démontré, par des essais très encadrés, la pertinence du traitement proposé ! Le souhait du Gouvernement n'est pas d'interdire le dépistage prénatal des pathologies pour lesquelles nous avons un système fiable

L'IMG est proposée lorsque la poursuite de la grossesse fait courir un risque grave à la mère ou lorsque le foetus présente un grave handicap physique ou mental, rendant son existence difficile ou sa survie impossible. Il s'agit d'une opération douloureuse. Lorsque les futurs parents sont confrontés à une suspicion de handicap de leur enfant, la réaction la plus naturelle est l'effet de panique. Sous le choc de l'annonce du diagnostic, ils ne sont pas forcément en mesure de l'assimiler. C'est pourquoi le délai de sept jours, qui est théoriquement prévu, est réellement important. C'est un temps de réflexion, de questionnement, de compréhension de la situation, ainsi que d'accompagnement. Ce délai de sept jours humanise tout simplement la démarche que s'apprête à faire le couple. Le Conseil d'État a lui-même considéré que ce délai était un droit important. L'inscrire dans la loi renforce ce droit. Par ailleurs, supprimer la proposition de ce délai de réflexion d'une semaine conduit à banaliser un acte qui a de lourdes conséquences humaines et psychologiques au détriment des alternatives que constituent l'accueil et la prise en charge des nouveau-nés malades ou handicapés. J'insiste sur le fait que ce délai de réflexion est une proposition faite aux femmes, aucunement une obligation. L'objet de cet amendement est d'accorder un droit à la femme, dont elle pourrait disposer si elle le souhaite.

long. Il nécessite une première phase de réalisation d'examens complémentaires afin d'évaluer le pronostic d'une pathologie particulièrement grave chez un foetus présentant une anomalie. ensuite le temps du diagnostic, le temps de l'annonce et des explications qui sont délivrées par l'équipe du centre à la femme ou au couple,

couples. De fait, une fois actée la décision de la femme, l'organisation de la prise en charge exige un temps de préparation incompressible.

La décision prise est le point d'aboutissement d'un très long processus qui demande beaucoup de confiance et d'échanges entre l'équipe médicale et le couple ou la femme qui prend cette décision. Rajouter un délai

ayant appris tous les dangers que fait encourir la grossesse telle qu'elle se présente, n'a qu'une seule solution véritable, celle d'interrompre la grossesse du point de vue médical.

Lorsque la difficulté est confirmée et que le risque est patent pour l'enfant ou pour la mère, et que le médecin et l'équipe médicale,

à partir du dépistage d'une anomalie entraînant des examens complémentaires ? À partir du moment où tous les examens complémentaires ont été confirmés ? À partir de celui où la femme, ou le couple, revient voir le médecin pour lui annoncer sa décision ? Et là, on leur dirait : « Votre décision est prise ?

à supprimer la clause de conscience inscrite dans le texte en cas d'interruption médicale de grossesse. Nous avions d'ailleurs déposé le même amendement en commission, mais celui du rapporteur était plus complet et mieux rédigé- c'est normal, c'est le rapporteur notamment sur l'obligation d'informer la patiente du refus du praticien et de lui communiquer le nom d'un collègue volontaire. Comme d'autres, je pense que cette double clause de conscience, spécialement pour les IMG, comme d'ailleurs pour les IVG, est inutile et superfétatoire. Nous avons déjà eu ce débat dans l'hémicycle. Une clause de conscience générale existe déjà pour tout médecin, comme comme pour les sages-femmes, pour tout acte médical. Pourquoi traiter l'IVG et I'IMG à part ? Je ne peux m'empêcher de penser, mes chers collègues, qu'il s'agit bien là, au XXI siècle, de continuer à vouloir contrôler le corps des femmes.

de cette double clause de conscience et mesurer son éventuel impact dans l'accès aux soins. Très sensible à cette question, elle nous avait dit lors d'un précédent débat qu'elle allait recevoir cette évaluation et nous la communiquer. Je vous remercie, par avance,

M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement a pour but de rétablir la clause de conscience spécifique pour l'interruption médicale de grossesse dans les termes votés par l'Assemblée nationale. En droit actuel, les médecins, sages-femmes, infirmiers et auxiliaires médicaux ne sont pas tenus de pratiquer une IMG, ou même seulement d'y concourir. Par souci de lisibilité du droit, l'Assemblée nationale a réécrit l'article pour énoncer explicitement les dispositions de la clause de conscience. membres de la commission spéciale du Sénat ont pu penser, étant donné que seul un médecin peut pratiquer une IMG, que lui seul était concerné par la clause de conscience et qu'il convenait ainsi de supprimer les dispositions relatives aux sages-femmes, infirmiers et auxiliaires médicaux. Or cela est inexact car, même si ces derniers ne peuvent en effet pratiquer eux-mêmes l'IMG, ils peuvent être sollicités pour y concourir. Supprimer cette clause de conscience est donc une régression par rapport au texte de l'Assemblée nationale et par rapport à l'état actuel du droit. Les débats qui ont eu lieu depuis plusieurs jours au Sénat montrent combien la confrontation à la maladie d'un enfant à naître ne reçoit pas de réponse univoque, combien elle entraîne un choix difficile et de nombreuses questions. Les auxiliaires médicaux sont confrontés à ces difficultés au quotidien. Les difficultés que rencontrent les professionnels de santé concernés pour faire valoir et respecter leurs choix éthiques montrent qu'en cette matière, on ne peut se contenter de faire valoir une clause de conscience générale. Mes chers collègues, il est important de protéger la liberté de conscience, surtout dans le contexte actuel d'offensive contre la liberté de conscience des personnels de santé. Il est donc impératif de rappeler, dans les dispositions du code de la santé publique relatives à l'IMG, la possibilité pour les auxiliaires médicaux

La commission spéciale a acté le fait qu'une clause de conscience générale permettant déjà de ne pas accomplir un acte contraire à ses convictions bénéficie aux professionnels de santé intervenant dans les dans les procédures d'interruption médicale de grossesse. Cette clause de conscience générale est aujourd'hui inscrite à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique qui prévoit que, « hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles ». Il s'agit bien d'une clause de conscience générale, laquelle permet à tout praticien de refuser des soins qui heurteraient ses convictions personnelles. Dans un rapport de 2011, le Conseil national de l'ordre des médecins, dont je rappelle qu'il est l'institution chargée du respect de la déontologie des médecins,

dans la requête qu'il a entreprise. » Aujourd'hui, le droit en vigueur en matière d'interruption médicale de grossesse renvoie donc aux dispositions applicables en matière de clause de conscience. L'absence de clause de conscience spécifique pour l'IMG n'a donc jamais empêché un médecin de refuser de pratiquer une IMG, le praticien pouvant se fonder sur la clause de conscience générale. Par ailleurs, au début de l'examen de ce texte, une clause de conscience spécifique avait également été proposée pour les médecins réalisant des actes de procréation médicalement assistée. Pour les mêmes raisons, notre assemblée avait décidé de repousser cette clause de conscience spécifique. Enfin, j'ajoute que la multiplication des clauses de conscience spécifique, qui n'a aucune portée en droit et n'aurait aucun intérêt, risquerait même d'affaiblir la clause de conscience générale. L'avis est donc défavorable. Quel est

En effet, l'article 21 du projet de loi présenté par le Gouvernement a pour but de supprimer le jeu de renvoi qui existe actuellement dans le code de la santé publique en matière de clause de conscience et de consentement des mineurs, car ce renvoi crée des confusions. Par exemple, les équipes des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal, confrontées à des interruptions de grossesses chez les mineures souhaitant garder le secret à l'égard de leurs parents, se sont interrogées à plusieurs reprises sur la position à adopter et les textes à appliquer. Par un effet de parallélisme, nous avons donc souhaité que cet article ne ne crée pas une nouvelle clause de conscience, mais que la clause de conscience applicable à l'IMG reste la même que celle applicable actuellement à l'IVG.

d'éviter toute confusion. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote. Je m'apprêtais à dire à M. Chevrollier que le groupe socialiste ne voterait pas son amendement, ce dont il se doutait doutait ... Notre collègue rapporteur Bernard Jomier a très bien répondu sur le caractère superfétatoire de la clause de conscience. Mais, d'un certain point de vue, je reconnais à M. Chevrollier une cohérence dans les amendements qu'il dépose. Il s'agit tout de même de sortir l'IVG et l'IMG des actes médicaux que pratiquent les médecins, déjà soumis à une clause de conscience contenue dans le code de déontologie, pour en faire des actes à part, dans le but à la fois de compliquer l'accès à ces actes, de culpabiliser les femmes

vous réaffirmez l'idée selon laquelle le code de déontologie ne suffirait pas à accorder à chaque soignant une clause de conscience générale, et que l'IVG et l'IMG seraient des actes médicaux à part qui heurteraient la conscience des médecins. Je note, en me

Je ne ferai pas davantage de commentaires, car je trouve que nous avons eu, depuis une dizaine de jours, un débat serein, apaisé et digne. Je ne souhaite donc pas tomber dans une certaine forme de provocation. Je voterai l'amendement défendu par M. Chevrollier pour les raisons qu'il a invoquées et pour celles que le Gouvernement, par le truchement de Mme la ministre, a exposées. Je le voterai aussi pour une autre raison, madame Rossignol : pendant ces dix jours de débat, nous avons tous fait montre d'un grand respect des opinions des uns et des autres.

second. Si, dans ce pays, on est incapable de respecter la liberté de conscience et la liberté de croire de chacun, l'intolérance est au bout du chemin. C'est extrêmement clair : je voterai cet amendement.

Sincèrement, je ne comprends pas que l'un de nos collègues se permette d'arriver en milieu d'après-midi pour enflammer l'hémicycle en donnant des leçons de morale, de raison et d'intelligence. J'assume, comme chacun de nous, ce que je pense, tout en sachant que je ne détiens pas la vérité- je n'aurai pas cette prétention.

nous devons être exemplaires en matière de respect des opinions et de démocratie. Très bien ! Certains propos qui ont été tenus dans cet hémicycle ne sont pas dignes et ne relèvent pas du tout d'un esprit démocratique et respectueux des opinions.

il soit là encore procédé, de manière affichée et inutile juridiquement- car je ne fais que du droit -, à une restriction de l'accès à l'IMG. Voilà ce qui me gêne.

les positions de ceux qui ne partagent pas les miennes. C'est ce qui fait la grandeur du débat parlementaire et qui doit aussi faire celle du débat public dans notre pays.

La clause de conscience du médecin est, me semble-t-il, importante, et il faut absolument la respecter dans tous les cas. Mais, à partir du moment où il accepte de faire cet acte d'IMG, il faut absolument qu'il puisse être

Mes collègues ont déjà à plusieurs reprises relu l'alinéa 10 de l'article 21, qui prévoit le cas du refus.

-le parallélisme qu'elle a fait entre l'IVG et l'IMG. L'IVG, c'est une interruption « volontaire » de grossesse. La clause de conscience spécifique pour l'IVG a été mise en place pour les raisons que vous connaissez et sur lesquelles je ne vais pas revenir. L'IMG, c'est une interruption non

la clause de conscience générale existe dans le code de déontologie des médecins, ainsi que dans le code de déontologie des autres professionnels de santé qui ont un ordre, en particulier les infirmiers.

qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer sans délai l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention ». Non seulement la clause de conscience existe dans les codes de déontologie des différentes professions médicales concernées par le sujet, mais en plus elle figure aussi dans le texte puisque nous l'avons prévue à l'article 21 ! La parole est à Mme la ministre.

l'article 21 a pour objet de clarifier les conditions de ce qu'on appelle une IMG pour les mineures. Qu'est-ce qu'une IMG ? C'est une interruption volontaire de grossesse pratiquée pour motif médical.

Il nous paraît donc important, par souci de parallélisme, de garder la clause de conscience prévue dans les cas d'IVG à moins de douze semaines,

la situation est différente. Il n'y a pas le même débat autour de la légitimité de la pratique de l'IMG : je n'ai entendu personne, sur aucune remettre en cause le droit d'une femme à pratiquer une IMG, qui est une procédure particulièrement douloureuse et pénible. Le parallélisme politique des formes ne s'applique donc

je prends l'exemple du secret médical, nous estimons que ce code prévaut : le secret médical protège le patient. Nous ne voulons pas ouvrir de brèche : on ne peut donc pas dire qu'on va se servir de notre code de déontologie à certains moments et pas à d'autres. Madame la ministre, je n'ai vraiment pas compris ce que vous disiez. Je pense que notre code de déontologie nous permet de ne pas effectuer cet acte si on y est opposé. Je suis vraiment de l'avis de mes confrères et je voterai contre cet amendement.

informer réellement les familles, sans évoquer, bien sûr les conséquences sur la vie de l'enfant et sans chercher de réel consentement. Imaginez, mes chers collègues, le désarroi des parents soumis, dans ce moment difficile, à une double pression : celle de l'appréhension binaire de notre société de l'injonction à déclarer le sexe administratif de leur enfant. L'orientation systématique vers les centres de référence spécialisés est déjà, pour nous, essentielle ; cela permet de garantir une prise en charge adaptée par des équipes pluridisciplinaires et d'instaurer, pour les cas les plus complexes, un échange avec les familles et les enfants avant toute intervention, si l'urgence vitale le nécessite.

rappelle, hors motif médical d'urgence vitale, « il convient d'attendre que le mineur soit en état de participer à la décision, et notamment de faire état de la souffrance qu'il associe à sa lésion et de moduler lui-même la balance avantage-risque de l'acte envisagé ». Il s'agit ainsi de ne plus laisser le monopole de la décision aux seuls médecins, de donner à l'enfant le temps d'être en mesure d'exprimer sa volonté et de participer à la prise de décision le concernant. un équilibre fragile entre un principe de non-interdiction, visant à laisser la capacité aux équipes médicales d'appréhender la nécessité d'une intervention, et la volonté de prévenir le recours systématique à la chirurgie précoce en l'absence d'une urgence vitale. Les travaux de ma collègue Maryvonne Blondin rejoignent les conclusions des rapports internationaux et la convention internationale des droits de l'homme.

que les souffrances des uns et les pratiques des autres soient respectées et que de nouvelles pistes de prise en charge soient élaborées pour l'avenir. Ainsi, en droite ligne de la recommandation que le Comité national d'éthique a formulée au travers de la commission a choisi de soumettre le diagnostic et la prise en charge de ces enfants à des recommandations de bonnes pratiques arrêtées par la Haute Autorité de santé. Pourquoi ?

termes du code de déontologie médicale, « aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement Malheureusement, cette partie du code ne nous semble pas toujours appliquée, notamment pour les 1,7 % d'enfants qui naissent, en France avec une variation du développement sexuel.

On ne peut que s'en réjouir, me semble-t-il, car comment peut-on imposer arbitrairement à des enfants des choix aussi binaires que le masculin ou le féminin, avec le risque que, quelques années plus tard, ce sexe ne corresponde pas

avec, évidemment, des dérogations : en cas d'urgence vitale ou de consentement explicitement et personnellement exprimé par la personne, même mineure. Ces opérations constituent une violence infligée à des personnes et elles ont des effets secondaires

de consentement personnel du patient mineur, lorsque celui-ci a suffisamment de discernement. L'adoption de ces amendements limiterait les opérations précoces pratiquées sur les enfants présentant des variations du développement génital aux seuls cas d'urgence ou de nécessité vitale.

du dissensus au consensus ». C'est dans cet esprit que la commission spéciale a adopté la disposition relative aux recommandations de bonnes pratiques,

Enfin, je note que l'adoption de l'amendement n° 61 rectifié ferait disparaître une disposition du code de la santé publique qu'il paraît important de conserver : la possibilité, pour un médecin, de délivrer les soins indispensables sur un mineur ou un majeur sous tutelle, malgré l'opposition de la personne titulaire de l'autorité parentale

ce sujet : « Hors motif médical très sérieux, il convient d'attendre que le mineur soit en état de participer à la décision, et notamment de faire état de la souffrance qu'il associe à sa lésion et de moduler lui-même la balance avantage-risque de l'acte envisagé. [ L'acte médical ayant pour seule finalité de conformer l'apparence esthétique des organes génitaux aux représentations du masculin et du féminin afin de favoriser le développement psychologique et social de l'enfant ne devrait pas pouvoir être effectué tant que l'intéressé n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté et de participer à la prise de décision.

En effet, dans certains types de cancers du sang, les lymphocytes T sont prélevés, cryopréservés, puis modifiés génétiquement afin de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses, avant d'être réinjectés au patient. La qualité des cellules prélevées et sélectionnées en amont joue un rôle important dans la faisabilité et la qualité du lot de cellules produit. Or le prélèvement et la cryopréservation ne sont actuellement réalisés que tardivement dans l'avancement de la maladie, entraînant une possible altération

notamment à une recommandation du récent symposium international sur les cellules, organisé par la faculté de médecine de Lille.

en améliorant la « qualité » du prélèvement initial des lymphocytes T, en vue de l'obtention de cellules. Le postulat de l'amendement est que ce prélèvement intervient aujourd'hui de manière trop tardive. Or dispose-t-on d'études médicales justifiant de l'intérêt d'un tel prélèvement de précaution avant les traitements de première intention ? D'après l'ANSM, aucune demande de clinicien souhaitant faire conserver les cellules de leurs patients en amont de l'administration des premiers traitements ne lui serait parvenue à ce jour. Si tel était le cas, en effet se demander si le cadre juridique actuel ferait obstacle à cette possibilité au point de justifier une intervention du législateur. L'article L. 1241-1 du code de la santé publique encadre le prélèvement de tissus ou de cellules « en vue de don », en précisant que cela ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un prélèvement « en vue de don », est-ce que ce cadre pourrait s'avérer trop restrictif ? En raison des questions soulevées, la commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement

Cette proposition est justifiée par le fait que ce type de traitement innovant intervient généralement après d'autres lignes de traitement, lesquelles ont pu altérer les cellules du patient. Dans ce contexte, elle s'inspire de ce qui est prévu pour l'autoconservation des gamètes, lorsque des traitements susceptibles d'altérer la fertilité sont mis en oeuvre.

D'un point de vue scientifique, je ne suis pas certaine de l'intérêt de prélever des cellules en phase précoce d'une maladie maligne, et ce pour plusieurs raisons. L'une des prochaines indications envisagées pour les est, par exemple, le myélome. Or, dans cette maladie, il y a lymphopénie, c'est-à-dire un très faible nombre de lymphocytes T. On le voit bien, dans ce cas-là, un prélèvement précoce poserait question. En outre, la technique utilisée aujourd'hui pour le prélèvement de ces cellules pourrait s'avérer inopérante avec la technique qui sera utilisée demain, car nous sommes en pleine phase d'expansion de la recherche ; la production des évolue en permanence, et les cellules prélevées pourraient finalement ne pas l'avoir été correctement ou ne pas trouver de finalité thérapeutique. telle disposition conduirait à des prélèvements conservatoires pour tout un tas de pathologies, sans tenir compte de l'impact organisationnel important que cela aurait, alors que la finalité thérapeutique pour le patient ne peut pas être avérée au moment du prélèvement. Enfin, cela a été dit par le rapporteur, l'article L. 1241-1 du code de la santé publique conditionne le prélèvement des tissus ou des cellules à une finalité avérée. Cela signifie que les dispositions législatives actuelles n'empêchent, à ce jour, ni le prélèvement ni la conservation de cellules d'un patient, si le protocole thérapeutique est dûment justifié et accepté par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), lors de l'évaluation du dossier d'autorisation de médicaments de thérapie innovante préparée pour le patient.

à modifier la paroi des lymphocytes T, de façon à ce que ceux-ci reconnaissent les cellules cancéreuses et les tuent.

ils ont vraiment besoin que des choses se mettent en place pour pouvoir avancer plus avant dans ces traitements, qui sont quand même très favorables aux patients. Il ne s'agit bien sûr pas de le faire en première intention, mais, pour ces traitements, ils ont besoin de lymphocytes T dans le

? Je me rangerai plutôt à l'avis du Gouvernement. Effectivement, il semblerait que, à l'heure actuelle, rien n'indique que la technique doive être modifiée. Cela dit, je ne

un très grand intérêt thérapeutique. Des greffes à partir de sang de cordon peuvent être envisagées, en particulier pour les maladies du sang.

En rendant possible la conservation de sang de cordon au sein de « banques », cet amendement reviendrait sur le caractère anonyme et gratuit du don, qui encadre aujourd'hui le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire.

rappelle qu'« il n'y a actuellement aucune preuve de l'efficacité et de la sécurité d'une telle utilisation autologue dans le traitement des maladies malignes ». Elle considère par exemple que la transplantation de sang de cordon autologue n'apporte pas les cellules immunitaires capables d'éliminer les cellules leucémiques,

Cette technique consiste à utiliser des virus mangeurs de bactéries présents en quantité abondante dans la nature ou le corps humain, les phages, afin de traiter certaines infections multirésistantes aux antibiotiques. Dans un contexte où l'antibiorésistance constitue constitue une des plus graves menaces, selon l'Organisation mondiale de la santé, nous devons donner toute sa place à la phagothérapie dans notre arsenal de soins pour traiter des patients qui se trouvent dans une impasse thérapeutique et, trop souvent, en phase finale. Cette technique, découverte par le professeur Félix d'Hérelle en 1917, est tombée en désuétude après la découverte de la pénicilline. Elle est toujours en vigueur dans les pays de l'ex-URSS, tels que la Géorgie, ou la Pologne, ce qui entraîne actuellement un tourisme médical de la part de patients pour lesquels pour lesquels les antibiotiques ne sont plus efficaces. Toutefois, ce dernier est réservé à ceux qui peuvent le financer, pour obtenir des bactériophages adaptés à leur infection. Les exemples de réussite se multiplient ! Je rappelle que la prise de phages n'a pas d'effets secondaires : cela marche ou pas, sans aucune autre conséquence. Je salue le travail en cours en cours d'une chercheure de Roscoff sur les phages d'origine marine. Pourquoi faut-il avoir recours, en France, à l'ATU ? Parce que les normes de production des phages sont plus strictes, et c'est normal, que celles d'autres pays. Des essais précliniques et cliniques ont été faits,

CSST, c'est-à-dire des comités scientifiques spécialisés temporaires, ont été mis en place dès 2016 par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Le dernier, de mars 2019, corrèle l'élargissement de l'accès aux bactériophages aux standards de qualité de la production industrielle. Or il faut savoir Or il faut savoir que l'industrie pharmaceutique n'est pas proactive à se saisir des produits naturels, vivants et non brevetables. Le CSST plaide pour la mise en place d'une plateforme nationale d'orientation et de validation du recours aux phages. J'espère, madame la ministre, qu'un coup d'accélérateur sera donné à cette demande, qui vient compléter le panel de la lutte contre l'antibiorésistance. La parole

tant au stade des essais cliniques que du don habituel pour une utilisation des selles à des fins thérapeutiques. Le niveau de contraintes imposé au donneur est très élevé du fait de la nature même du don et des étapes nécessaires pour la qualification d'un donneur. En effet, le candidat donneur accepte de subir des examens médicaux répétés, des tests sanguins et des tests de selles, le tout selon les règles de sélection biologique et clinique applicables. Il s'engage aussi à faire des dons réguliers, en général quotidiens. Dans ce contexte, seuls 3 % des candidats sont qualifiés. Que les dons soient réalisés sur place, amenés au centre ou collectés par un coursier, le process de collecte influe sur l'organisation personnelle, pouvant impliquer des impacts financiers. Le donneur s'engage également à respecter une hygiène de vie, notamment concernant son alimentation, pendant la durée de la collecte. Il en est de même pour les donneurs retenus au terme de ce processus de sélection, qui se prêtent de façon habituelle au don de selles et dont les frais doivent pouvoir être pris en charge par les établissements et organismes autorisés. Cet amendement peut paraître incongru-

: La parole est à Mme Michelle Gréaume. Par cet amendement, nous proposons d'élargir la composition du Comité consultatif national d'éthique aux représentants des associations directement concernées par les questions de bioéthique. Nous considérons en effet que la bioéthique n'est pas seulement une affaire de sachants, même si nous ne remettons bien entendu pas en cause la compétence et les apports importants des experts, qu'ils soient médecins, chercheurs ou encore juristes, lesquels occupent une place légitime au sein du CCNE. Les questions de bioéthique prennent de plus en plus de place dans le débat public et suscitent un intérêt croissant chez nos concitoyens, y compris chez les plus jeunes. Nous devons saluer et encourager

La discussion sur les enjeux majeurs qui sont devant nous doit pouvoir s'appuyer sur ce triangle que j'évoquais entre parlementaires, experts et citoyens. Il s'agit d'une construction commune. La santé se prête bien à ce type de discussion. Par ailleurs, le CCNE, dans son avis sur la révision de la loi Bioéthique 2018-2019 et fort de l'expérience des États généraux de la bioéthique, a appelé de ses voeux une intensification de la participation de la société civile dans les débats relatifs à la bioéthique. C'est le sens de cet amendement, qui vise à élargir la composition du CCNE à six représentants d'associations de personnes malades et d'usagers du système de santé,

Même si elle n'est pas expressément prévue, la présence au sein des membres du CCNE de représentants du monde associatif est possible, notamment au sein du collège des personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique. Le CCNE comprend ainsi aujourd'hui la présidente

impliquant les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites, introduites au V de l'article L. 2151-6 et au V de l'article L. 2151-7

auteur. Le sujet est le régime d'autorisation des recherches conduisant à la création d'embryons chimériques par insertion dans un embryon animal de cellules souches embryonnaires ou pluripotentes induites humaines. Depuis la suppression

Finalement, il aura fallu trois jours la semaine dernière et deux cette semaine. Cela est évidemment dû à la grande sagesse des sénateurs,

Je voudrais donc vous remercier, mes chers collègues, de ce travail important et intéressant. Je voudrais aussi remercier les

que nous sommes nombreux à nous interroger sur l'équilibre du texte, tel qu'il a été modifié par le Sénat. Chacun avait probablement en tête son texte idéal ; aucun ne le retrouvera sans doute dans le texte adopté,

accueillir les innovations, les mettre au service des patients, dans le respect de nos principes éthiques. Qu'a adopté le Sénat ? Je vais citer quelques points saillants, sans revenir sur tous les articles l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, mais en conservant les principes qui régissent le médical et le sociétal ; un mode d'établissement de la filiation qui respecte, là encore, nos principes un accès aux origines qui fait droit aux demandes qui s'expriment aujourd'hui, c'est-à-dire celles des enfants déjà nés de dons, qui étaient écartées du texte

Le Sénat a modifié le régime d'autorisation de la recherche sur l'embryon, interdit les chimères, rétabli le DPI-HLA, mais a refusé d'accepter d'autres dépistages, tout comme les tests généalogiques.

Agnès Buzyn et Nicole Belloubet, ainsi que de l'ensemble de nos collaborateurs, de vous remercier de ce temps de travail que nous avons passé ensemble. C'est toujours un moment extrêmement enrichissant, surtout sur des questions comme celles que nous avons abordées dans ce projet de loi de bioéthique,

de savoir ce que la science permet, certes, mais, surtout, ce que nous souhaitons qu'elle apporte à la société. Parfois, ce que la science permet n'est pas toujours souhaitable dans une société. Nous n'avons pas été d'accord sur tout, bien sûr. sûr. Quoi qu'il en soit, les débats ont toujours été de très grande qualité. Je voulais adresser mes remerciements tout particulièrement à la commission spéciale et aux rapporteurs,

je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public sur l'ensemble du texte se dérouleront le mardi 4 février, à